sur les conclusions du rapport d'information. Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses, dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, aucune technologie ne peut être neutre, car toutes portent en elles une vision du monde. La délégation à la prospective du Sénat a réfléchi, à la demande de son président, M. Roger Karoutchi, à la question de l'impact sur l'emploi de l'utilisation de plus en plus fréquente de robots et de machines intelligentes dans toutes les sphères d'activité, publiques ou privées. des robots n'est plus l'apanage de la seule industrie pour effectuer des tâches pénibles et répétitives. Nous voyons se déployer rapidement des systèmes automatiques qui réalisent mieux que nous des tâches qui nous étaient jusque-là imparties dans notre activité quotidienne. Certes, un monde où l'ensemble des tâches, des plus banales, comme conduire une voiture ou faire la cuisine, aux plus complexes, comme analyser une masse de documents, seraient effectuées par des machines, cela relève encore de la science-fiction. la révolution des robots est déjà là. Une technologie joue un rôle important dans ce vaste mouvement vers l'automatisation : l'intelligence artificielle, l'IA. Elle a connu un essor spectaculaire durant la dernière décennie, avec le développement de l'apprentissage automatique ou les réseaux de neurones profonds.

L'impact de cette révolution technologique sur l'emploi inquiète. Les salariés peuvent-ils être remplacés par des machines ? Ce mouvement a déjà été observé de manière massive sur les chaînes de production industrielle. Il concerne aussi désormais les services : caisses automatiques, applications de recherche de vols et de voyages en ligne, analyse de la solvabilité des emprunteurs par les banques Les services ne sont donc pas épargnés par le mouvement d'automatisation des tâches. Or les emplois de service représentent 75 % de l'emploi en France. Même des métiers qualifiés sont touchés : le radiologue est désormais en concurrence avec la machine pour lire avec précision un cliché radiographique, les des salles de marché sont remplacés par des ordinateurs effectuant du à haute fréquence. Le rapport Frey-Osborne de 2013 estimait que 50 % des emplois risquaient de disparaître aux États-Unis en vingt ans, sous l'effet de l'automatisation des tâches. Les estimations plus récentes sont moins effrayantes des travaux laissent penser que seulement de 10 % à 15 % des emplois existants aujourd'hui sont menacés de disparition du fait de l'automatisation. Des compensations paraissent donc possibles au niveau macroéconomique, avec la création d'emplois pour exécuter des tâches non automatisables. émerger un chômage technologique de masse ne nous paraît donc pas fondée. Cette hypothèse ne s'est jamais vérifiée dans l'histoire. Les pays les plus robotisés, comme l'Allemagne, le Japon ou la Corée du Sud, sont aussi ceux qui ont le taux de chômage le plus faible. En revanche, les experts ont une certitude : de très nombreux emplois vont être transformés par l'automatisation. Les compétences attendues des salariés, l'organisation du travail risquent d'être bouleversées assez rapidement par un progrès technologique rapide. Il ne faut pas croire que, par nature, certaines activités seront épargnées. Nous avons observé que, dans de nombreux domaines- l'agriculture, la logistique et les transports, la sécurité et la défense, les services financiers, le commerce, les loisirs, l'énergie, l'environnement, les services juridiques et même le soin et l'accompagnement des personnes âgées -, les robots les robots se diffusent, parfois pour améliorer l'efficacité du travail humain, mais parfois aussi pour le remplacer en automatisant des tâches. Dans les transports, la perspective du véhicule autonome conduit à envisager la fin des métiers de chauffeur routier ou de taxi. Ne croyons pas non plus que des services à forte dimension relationnelle ne soient pas automatisables, au moins en partie : l'accueil dans les hôtels ou l'animation d'un atelier dans une maison de retraite peut être confié à un robot, une procédure administrative peut être remplacée par une téléprocédure. Le plus grand risque d'automatisation pèse personnels administratifs gèrent des procédures assez normées facilement exécutables par des machines. Leur savoir-faire, une fois « encapsulé » dans des algorithmes, ne leur appartient plus et se trouve transféré aux machines. De tels salariés sont appelés à évoluer rapidement vers des tâches nouvelles, qui ne sont pas confiées à des machines pour des raisons techniques ou économiques, faute de quoi ils perdront leur emploi. Tout est plus incertain, et une question fondamentale nous est posée : sera-t-on capable de répondre à ce besoin d'adaptation ? Ne versons pas dans le pessimisme, et préparons-nous à ce changement, préparons-nous à une robotisation heureuse !

Madame la présidente, monsieur le président de la délégation, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de Mme Agnès Pannier-Runacher et de M. Cédric O, retenus par d'autres engagements. Je voudrais tout d'abord revenir sur le constat fait par la délégation sénatoriale à la prospective et partagé par le Gouvernement : les besoins de main-d'oeuvre liés à la révolution numérique sont massifs, notamment dans les domaines du social, de la mobilité, de l'analyse des données, des services, du ou de la sécurité. Selon la Commission européenne, 756 000 postes sont à pourvoir par des experts du numérique en 2020, dont 212 000 en France. selon Syntec Numérique, syndicat de l'industrie du numérique, il existe un déficit annuel de 10 000 diplômés dans ce domaine. La révolution numérique implique des transformations globales, tant du marché du travail, puisque 50 % des emplois sont ou seront concernés par cette transformation technologique, que de notre manière de former et de penser.

Un Capes « numérique » verra le jour en 2020. S'agissant de l'accès aux opportunités économiques offertes par la révolution numérique, le programme French Tech Tremplin a été mis en place. Doté de 15 millions d'euros, il a pour objectif d'aider les porteurs de projet éloignés de la technologie- demandeurs d'emploi, jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, etc. -à créer leur entreprise ou à en accélérer le développement. Les lauréats bénéficieront d'une bourse, d'un parcours d'accompagnement et d'un soutien rapproché et personnalisé de la part d'un mentor.

Pour des raisons de compétitivité, les entreprises françaises devront à terme s'approprier et intégrer les technologies de l'intelligence artificielle. Cette appropriation se concrétisera par le recrutement de spécialistes hautement qualifiés, hautement qualifiés, mais également par la diffusion d'une formation à l'intelligence artificielle à tous les échelons de l'entreprise. La formation à l'intelligence artificielle est un enjeu majeur, comme l'a justement souligné le rapport de la délégation. En matière de formation de spécialistes, par exemple de, l'écosystème éducatif français est mondialement réputé. Structuré, il se développe notamment grâce au volet « expertise » de la stratégie nationale de l'intelligence artificielle déployée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ainsi, de multiples mastères spécialisés en intelligence artificielle existent en France. Concernant la formation et la sensibilisation à l'intelligence artificielle à destination des professionnels non spécialistes, le champ reste encore peu couvert. Cependant, plusieurs actions françaises et européennes ont été entreprises, notamment par l'intermédiaire de (MOOC), sur l'initiative de l'université

au travers des et de l'intelligence artificielle. Elle est le fruit d'une recherche permanente d'innovations des acteurs du tourisme pour répondre aux besoins de clients, notamment étrangers, qui ont souvent besoin d'un accompagnement avant et pendant leur séjour dans leurs différentes démarches. Elle permet une réponse en temps réel, 24 heures sur 24 et dans toutes les langues, qui ne pourrait pas être assurée par des emplois physiques, améliorant ainsi la qualité du service aux touristes, leur expérience en France et, finalement, l'attractivité de la France en ce domaine. Elle n'a, dans ce cas, pas remplacé d'emplois physiques ; elle a surtout permis d'améliorer la relation clients. Le Gouvernement a encouragé, comme le préconise le rapport de la délégation, ce développement d'innovations par la mise en des données publiques sur le tourisme produites par les collectivités territoriales, la mise en place de la plateforme datatourisme.gouv.fr, il y a deux ans.

les automates et l'automatisation d'entrepôts peuvent permettre des gains de productivité, de temps, et être sources d'utilité économique, puisque le consommateur peut par exemple faire ses achats le dimanche, mais ils peuvent aussi induire un taux d'emploi plus faible, et donc de possibles restructurations. L'expérience montre toutefois que la part du recours à l'automatisation reste souvent mineure par rapport à celle de l'interaction avec des vendeurs, commerçants et caissières, à laquelle, je le crois, nous sommes tous attachés. Face à ces évolutions qui peuvent être contradictoires, le Gouvernement veille évidemment à ce que la robotisation ne permette pas de contourner le droit du travail. Le Gouvernement s'efforce en outre d'inciter les entreprises à accompagner leurs salariés vers des tâches à plus haute valeur ajoutée, afin que ceux-ci ne soient pas durablement exclus du marché du travail en raison de l'obsolescence de leurs compétences ou de leur métier. La question de l'impact du numérique sur l'emploi et les formations est primordiale ; il faut donc accompagner les différentes branches professionnelles pour former les travailleurs concernés. Je prendrai ici l'exemple des centres d'appel des entreprises, les, qui sont de plus en plus confrontés à la montée en puissance de la robotisation de la relation clients, laquelle permet de répondre aux demandes primaires des clients sans interaction

Ce secteur connaît un rythme de croissance annuelle de 3,5 %, avec un potentiel de création de 7 000 emplois par an. Concomitamment, l'intelligence artificielle et les pourraient conduire à la suppression de 7 000 emplois par an au cours des cinq prochaines années. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement a ouvert un chantier pour s'assurer que ce secteur pourra mobiliser tous les outils pour faire monter en compétences ses salariés 7 000 agents seront ainsi formés chaque année par la branche et l'opérateur de compétences du secteur. Comme le préconise le rapport sénatorial, le Gouvernement oeuvre donc à renforcer l'appareil de formation professionnelle en accordant une priorité aux travailleurs dont l'emploi est automatisé ou susceptible de l'être rapidement. En définitive, il me semble important de souligner la richesse que peut représenter la révolution numérique dès lors qu'elle est accompagnée par des femmes et des hommes : j'en veux pour preuve le secteur de la santé. Robotisation et numérisation offrent de très larges potentialités, qui devraient permettre d'apporter une réponse au déficit de personnel dans certains établissements et au domicile, mais cela nécessite d'importants investissements en termes de capital humain comme de capital technologique. Le déploiement d'assistants robotisés pourrait représenter une réelle opportunité en termes de réduction du coût du travail ou de gains de productivité. Ils peuvent apporter une présence 24 heures sur 24 et 7 jours je tiens à le préciser -d'une présence humaine dans les établissements et au domicile. Une politique importante de formation des personnels devra accompagner cette modernisation rapide des services. Des investissements pourraient en partie s'opérer grâce à la masse salariale non mobilisée du fait d'un déficit chronique de recrutement dans ces services avec des retours sur investissement rapides, de l'ordre d'un à deux ans. Des expériences françaises existent, qui pourraient, si l'on conclut à leur succès, être répliquées. Il convient toutefois de souligner que les activités de service à la personne, eu égard à la place centrale qu'y occupe le lien humain, ne se prêteront sans doute pas à une substitution très large du personnel par des robots, ce qui est heureux. Le Gouvernement est d'ailleurs bien plus attaché à la complémentarité de ces solutions qu'à leur opposition. L'État entend donc poursuivre son accompagnement d'initiatives dans ce domaine : il a lancé un projet d'concernant sa base de données sur les services à la personne, avec pour possible débouché la mise à disposition du public et des opérateurs des données anonymisées de la filière à relativement brève échéance. Ce projet rejoint en tout point la préoccupation du Sénat exprimée au travers de la recommandation n° 4 du rapport, concernant l'importance d'élaborer des politiques d'utilisation de la donnée publique et privée. Cette même prise en compte des femmes et des hommes salariés d'un secteur touché par la révolution numérique a également conduit le Gouvernement à mieux réguler l'activité des plateformes. La numérisation des différentes filières, notamment le développement rapide de plateformes, permet de dynamiser l'offre et de favoriser le fonctionnement d'un marché longtemps réservé réservé à quelques opérateurs. Le Gouvernement a lancé un chantier transverse sur l'émergence des plateformes et leur impact en termes de création de valeur et d'emplois. Des mesures de simplification de la réglementation existante seront proposées pour accompagner ce mouvement, notamment dans le secteur des services à la personne, où ces nouveaux acteurs renouvellent un modèle économique trop fragile, car les marges y sont trop faibles, mais également dans les domaines de la mobilité ou de la logistique, auxquels le rapport sénatorial fait à de à de multiples reprises référence. Un chantier doit par ailleurs être lancé, sur la base de l'habilitation que confère au Gouvernement l'article 48 de la loi d'orientation des mobilités, visant à clarifier et à encadrer la représentation des travailleurs au sein des sociétés de plateformes de services, afin notamment de refléter l'impact des nouvelles technologies de la donnée sur les conditions de travail.

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.

M. Roger Karoutchi. Monsieur le ministre, grandeur et servitude de la fonction : vous voilà maître des robots, en tout cas pour ce matin

et de sa place dans la société. Yann Le Cun, grand spécialiste français de l'intelligence artificielle, récent lauréat du prix Turing, nous dit qu'il « n'est pas sûr que la révolution de l'IA profite à tous Il estime que « tous les métiers sont concernés par ce changement » et que « l'IA rend plus précieux ce avec quoi elle ne peut rivaliser », ce qu'il appelle « l'expérience humaine authentique », faite d'émotion, de sensations, de relations humaines uniques, valorisée sur les marchés bien davantage

qui dilue toujours plus les classes moyennes, intermédiaires, pour ne laisser, d'un côté, que des acteurs productifs mobiles, et, de l'autre, des acteurs assujettis, des sédentaires au service de ces nomades créateurs de valeur.

gestation. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire par quelles politiques publiques à destination du plus grand nombre de nos concitoyens le Gouvernement appréhende ces bouleversements sociétaux et comment il compte associer les forces vives de la Nation- je pense aux corps intermédiaires et aux intellectuels, notamment -à

Ce secteur fait face à des difficultés importantes de recrutement, liées pour l'essentiel au manque d'attractivité des carrières. La faiblesse des rémunérations, la précarité, les fréquentes coupures dans la journée de travail et les nombreux déplacements sont souvent évoqués pour expliquer les pénuries de personnel. de personnel. En outre, les auxiliaires de vie peuvent être confrontés à des conditions de travail difficiles, avec des tâches traumatisantes pour le corps et, parfois, la violence physique et verbale de personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Au Japon, où la question du vieillissement de la population se fait encore plus prégnante, on estime qu'il manquera 370 000 soignants en 2025.

Pour l'heure, ces outils sont utilisés en maisons de retraite, mais on en voit déjà les applications possibles pour le maintien à domicile. Dans ce domaine, la domotique permet déjà d'améliorer le confort des personnes dépendantes et à mobilité réduite. Bien sûr, il n'est pas question de nier l'importance du lien humain, qui doit absolument être privilégié et préservé. Je sais d'ailleurs que l'attractivité des métiers de l'aide à domicile sera au coeur de la prochaine loi sur le grand âge et l'autonomie.

l'intelligence artificielle sont en train de bouleverser le marché du travail. L'OCDE annonce qu'un emploi sur six sera détruit par la numérisation de l'activité économique, et un sur trois substantiellement transformé. Ces chiffres peuvent faire peur, peur, mais ces technologies représentent aussi un véritable moteur de croissance et un gisement d'emplois potentiels : plus de 600 000 postes d'expert en numérique

faiblesses : fuite de nos cerveaux, rachat de nos jeunes pousses les plus performantes, notamment par de grands groupes américains. En vue de réussir notre adaptation, la Commission européenne a identifié un défi majeur : former un plus grand nombre de spécialistes en intelligence artificielle et créer un environnement de travail attractif pour enrayer la fuite des cerveaux. La Commission européenne envisage de consacrer chaque année 1 milliard d'euros à la recherche sur l'intelligence artificielle, ce qui devrait déboucher,

la compétitivité technologique de l'Union européenne, à anticiper les changements socioéconomiques et à créer un cadre juridique et éthique pour l'intelligence artificielle. Le programme Digital Europe, doté de 9,2 milliards d'euros, tend à renforcer les capacités numériques de l'Union européenne dans les supercalculateurs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les compétences numériques des citoyens. Le programme Horizon

La colère populaire se focalisa sur les machines, au motif qu'elles risquaient de priver les travailleurs de leur emploi. Depuis lors, nos économies se sont numérisées et mondialisées. Les données du problème ont radicalement changé, mais les mêmes craintes ressurgissent immanquablement. On craignait hier pour les emplois industriels ; on craint aujourd'hui pour les métiers des services. La robotisation va bien évidemment faire émerger de nouveaux emplois, mais d'autres seront voués à disparaître ou à évoluer. De nombreux économistes considèrent que la distinction stricte entre industrie et services est dépassée. Les deux secteurs deviennent de plus en plus indissociables. Plusieurs tendances sont à l'oeuvre, comme le développement de l'économie de la fonctionnalité, privilégiant la prestation d'un service à l'acquisition d'un bien, l'éclatement des chaînes de production entre une multitude d'acteurs ou encore la montée en puissance du travail intérimaire, considéré comme un service même lorsqu'il concerne la production industrielle. de compétitivité nous impose d'être à la pointe des développements technologiques. Cette mutation ne peut se faire sans un accompagnement individuel et la mise en place de formations adaptées pour les personnels concernés. Monsieur le ministre, comment le Gouvernement compte-t-il accompagner cette mutation ? Quelles mesures entend-il mettre en place pour soutenir la création d'emplois et, corolairement, compenser les pertes ? Quels sont les politiques et les leviers d'accompagnement de ces évolutions techniques et technologiques en matière d'emploi, de marché du travail, de droit du travail à

Pour l'année 2020, voici quelles sont nos pistes de travail. Le Président de la République a annoncé, en septembre, le lancement d'une gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences au niveau national, construite avec les régions, pour déterminer comment l'offre de formation devra évoluer en volume et en contenu dans les cinq à dix prochaines années. Cela renvoie aux propos de M. Karoutchi sur la nécessité de la prospective. Dans la foulée du Pacte productif, nous allons améliorer l'étude prospective des métiers et des qualifications, pour affiner encore la politique de formation et les outils d'orientation. Nous allons mobiliser le service public de l'emploi afin d'accompagner les start-up dans le recrutement des talents, avec l'appui des correspondants French Tech de Pôle emploi (APEC). Enfin, nous simplifions et rendons plus attractifs les outils d'intéressement au capital pour les salariés, aux fins d'attirer les jeunes talents dans les start-up et de compenser la faiblesse relative

prospective, Marie Mercier et René-Paul Savary, ont produit un passionnant rapport sur le thème « les robots demain », qui nous a permis, par la même occasion, de « démasquer » tous les robots d'aujourd'hui, du quotidien, ceux qui, parfois depuis hier, se sont discrètement et définitivement installés dans nos vies.

travail ». Or, comme vous tous ici, mes chers collègues, je suis un acteur impliqué de mon territoire, que je sillonne le plus souvent possible. Il me revient chaque jour que de très nombreux emplois ne sont pas pourvus, ce qui constitue parfois un frein au développement de services et d'activités industrielles et commerciales.

Je ne sais si cela passe par une forme de charte, d'éthique, de choix de politique publique, mais telle est, monsieur le ministre, la question que je voulais vous soumettre. J'ai par ailleurs les plus grandes réserves et inquiétudes quant à l'empreinte carbone de cette évolution.

À titre d'exemple, de manière provisoire, une baisse d'environ 9 % des emplois est envisagée dans le secteur de la finance et de l'assurance, mais, inversement, on s'attend à une hausse de 36 % des emplois dans les activités informatiques et de services. Enfin, le Pacte productif annoncé par le Président de la République vise à construire une gestion

existence : l'emploi, mais aussi nos modes de déplacement, nos loisirs, chacune de nos activités quotidiennes. Or, dans ce domaine, la France et l'Europe se sont laissé distancer par les États-Unis, forts de la puissance de frappe des Gafam, des Gafam, qui disposent d'un véritable trésor de guerre- les données de leurs utilisateurs, accumulées au fil des années -, et la Chine, qui, pour sa part, ambitionne de devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle à l'horizon de 2030. L'Europe dispose pourtant de tous les atouts pour rivaliser avec ces deux pays. Mais il faut agir vite ! Le nouveau commissaire européen français, M. Thierry Breton, a annoncé un plan pour une « politique européenne de la donnée

que l'intelligence artificielle fasse l'objet d'un projet important d'intérêt européen commun (PIIEC). Ce mécanisme permettrait à des États membres d'accorder au secteur crucial de l'intelligence artificielle des aides financières, en adaptant les règles de concurrence européennes. Cela serait bénéfique à l'ensemble de la société et de l'économie européennes, et donc à l'emploi.

Les acteurs économiques ont besoin de pouvoir accéder à des jeux de données importants, publics comme privés, pour déployer des solutions innovantes dans leurs processus de fabrication, ainsi que dans leurs produits et services. C'est un enjeu de compétitivité, et même de souveraineté. Cela a été dit, nous avons pris en la matière beaucoup de retard

Il est donc indispensable de favoriser la mutualisation des données, si l'on veut poursuivre le développement de solutions technologiques de pointe françaises et européennes autonomes. À l'échelon européen, la Commission a établi les lignes directrices visant à encourager l'ouverture des données privées à des fins d'intérêt public. Des plateformes comme Dawex constituent des exemples de réussite en la matière, démontrant largement la capacité des entreprises européennes à être compétitives dans ces secteurs. À ce titre, en matière d'économie de la donnée, la France et l'Union européenne se doivent de promouvoir et d'affirmer une approche respectueuse des droits de l'utilisateur. Cette approche constituera le socle de notre compétitivité de demain en matière de plateformes de partage de données. Néanmoins, il convient de garder à l'esprit que la production, le stockage et le traitement de données impliquent des contraintes de sécurité particulières, dont il est essentiel de faire cas pour faire émerger des plateformes de données européennes d'envergure mondiale. Il est donc désormais nécessaire d'arrêter une stratégie commune et opérationnelle pour jouer le rôle de catalyseur attendu de la puissance publique en matière de partage de données. Il convient notamment de s'interroger sur la nécessité de définir des typologies de données et des finalités d'accès claires en matière de politique industrielle et d'action publique, la définition d'un régime juridique encadrant les modalités d'ouverture, de partage et d'exploitation de ces données, la nécessité d'un recours à des tiers de confiance et le rôle des autorités de contrôle. À cet égard, des réflexions sont en cours, notamment au niveau européen, sur l'intérêt du partage de données

des emplois d'ici à 2025. Taxer les robots permettrait de freiner le remplacement du travail humain, donc de limiter le rythme des destructions d'emplois et, comme l'a dit Bill Gates, cité dans le rapport,

question. Elle permettrait aussi de redistribuer le revenu et de corriger les inégalités, car il n'échappe à personne que la richesse supplémentaire produite grâce à la robotisation du travail ne profite guère qu'aux actionnaires.

et a évoqué « l'éventuelle application d'un impôt sur le travail réalisé par des robots ou d'une redevance d'utilisation et d'entretien par robot. Cela devrait être examiné dans le contexte

Avant d'envisager de créer une nouvelle taxe, il faut s'attaquer au défi le plus urgent, à savoir augmenter le taux de robotisation dans notre pays. Il y va de notre souveraineté et de notre compétitivité. Ensuite, les obstacles juridiques sont nombreux. Pour appliquer une telle taxe, il faudrait déterminer avec précision son champ d'application, ce qui amènerait à établir une définition du robot et à fixer un seuil d'automatisation à partir duquel une machine serait considérée comme un robot. Un ordinateur et un logiciel pourraient-ils ainsi être considérés comme un robot ? De cette difficulté à définir les robots résulte non seulement une difficulté à déterminer la base imposable, mais aussi un sérieux problème de constitutionnalité. En effet, au regard du principe de l'égalité devant l'impôt, la détermination du champ d'application de la taxe doit être fondée sur des critères objectifs

d'ici 2025, les robots mettraient au tapis plus de 3 millions d'emplois dans l'Hexagone ». De plus en plus, ce n'est plus l'ordinateur qui assiste l'homme, mais l'homme qui assiste l'ordinateur. Aujourd'hui, comme hier, les robots alimentent les fantasmes les plus noirs, alors qu'ils ne font qu'ouvrir la voie à l'émergence de nouveaux métiers. En aout dernier, je faisais je faisais partie de la délégation française conduite par la ministre Muriel Pénicaud venue défendre à Kazan la candidature de Lyon à l'organisation des Olympiades des métiers en 2023, avec le soutien du Président de la République. les WorldSkills à Lyon en 2023 est une merveilleuse occasion de changer le regard porté par les Français sur l'apprentissage et la formation professionnelle. Nos compatriotes verront des jeunes de moins de 23 ans, venus du monde entier, en compétition dans soixante métiers artisanaux, industriels et numériques. Outre que ces olympiades des métiers donnent une image rafraichie et dynamique de métiers traditionnels, ils sont aussi une vitrine de la révolution numérique en cours, qui suscite constamment de nouveaux besoins, et donc de nouveaux métiers. Lors de la compétition à Kazan, Michel Guisemberg, président de WorldSkills France, et le comité qui l'entoure ont mis en évidence que, si la France était très bien représentée pour les métiers traditionnels, nous n'avions que peu de compétiteurs pour ces nouveaux métiers.

Vous avez raison, il faut accélérer, former plus et mieux aux métiers nouveaux liés à la révolution numérique. Je pense aux métiers de développeur, de ou d'intégrateur. Le Gouvernement est très actif en la matière, depuis l'école jusqu'à la formation continue.

pour déterminer l'offre de formation, qui devra évoluer en volume et en contenu dans les cinq à dix prochaines années. Nous oeuvrons actuellement avec le ministère du travail à la construction de plans d'action pour une sélection de métiers en tension prioritaires, ainsi que de propositions transverses pour améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande de compétences pour l'ensemble de l'économie. Il reste encore beaucoup à faire pour relever le défi du recrutement dans l'industrie numérique, qui est un formidable gisement d'emplois. Cela passe par la multiplication des forums

et la ligne 1, qui, elle, l'a été plus récemment, pour un montant de l'ordre de 629 millions d'euros. Monsieur le ministre, ma question est simple : le Gouvernement compte-t-il accompagner

est à Mme Viviane Artigalas. Les périodes de ruptures technologiques sont généralement marquées par des bouleversements majeurs de l'organisation du travail et suscitent dès lors de grandes inquiétudes. On se souvient du mouvement des luddites, au début du XIX siècle en Angleterre, ces ouvriers « briseurs de machines » qui cassaient les nouveaux métiers à tisser introduits par la révolution industrielle. Si la robotisation massive fait encore débat, l'effet des nouvelles technologies sur les conditions de travail n'est pas neutre. Je pense notamment à ces nouveaux travailleurs « ubérisés », devenus « servants » des machines numériques que sont les plateformes. À l'instar du taylorisme qui émiettait le travail, la révolution numérique risque, si l'on n'y prend garde, de le déshumaniser. comme toute révolution technologique, elle offre aussi de nouvelles opportunités pour améliorer considérablement les conditions de travail, notamment en diminuant la pénibilité de certains métiers. Cela suppose néanmoins une action des pouvoirs publics pour orienter les investissements en ce sens et encourager l'utilisation de ces nouvelles technologies dans nos PME et TPE, notamment celles du secteur des services, qui concentre des métiers particulièrement pénibles. Bien souvent, ces PME n'osent pas investir, eu égard à une rentabilité qu'elles jugent incertaine. Or il est indispensable que nos entreprises se modernisent et créent de nouveaux emplois qualifiés dans nos territoires. Monsieur le ministre, compte tenu de la nécessité d'une meilleure diffusion de la robotisation, le Gouvernement a-t-il prévu d'aider les PME et TPE du secteur des services, pour qu'elles ne ratent pas le coche de la modernisation et puissent recourir à des techniques permettant aussi d'améliorer les conditions de travail ?

de santé du travailleur et sur sa capacité à exercer son métier. Or la perspective de l'augmentation du taux d'emploi des seniors soulève la question de leur capacité à travailler plus longtemps. Parmi les principaux facteurs de pénibilité figurent le travail de nuit,

et des modifications dans les investissements des entreprises. Comme je l'ai déjà indiqué, le Gouvernement est pleinement investi sur le sujet de la formation, notamment pour développer des compétences dans le numérique. L'un des objectifs du Pacte productif est d'ailleurs d'atteindre le plein emploi en 2025. À cette fin, une étude prospective des métiers, des qualifications et des investissements nécessaires

au profit du plus grand nombre. Cela suppose, je le redis, de soutenir les PME en créant des aides spécifiques et en favorisant leur obtention. Monsieur le ministre, le Gouvernement ne doit pas faire la même erreur qu'avec l'article 41 de la loi d'orientation des mobilités, censuré par le Conseil constitutionnel, qui permettait aux plateformes numériques de définir elles-mêmes les caractéristiques essentielles du contrat de travail. de travail. Autrement dit, il ne faut pas laisser la main au marché et au privé pour réguler les relations de travail dans la nouvelle économie numérique ! Ce n'est pas de cette manière que l'on rassurera les populations qu'inquiète la rapidité des changements technologiques. Je reste cependant convaincue que, si l'on prend les mesures qui s'imposent pour canaliser les innovations, les nouvelles technologies peuvent être source d'amélioration et de progrès social au coeur de nos entreprises. La parole est à Mme Catherine Procaccia. En lisant les pages du rapport

de la population et à un manque de personnel soignant dans les hôpitaux et les maisons de retraite, le gouvernement japonais a massivement investi, dès 2013, dans des robots d'aide à la personne

Déclarer que les services à la personne sont une mine d'emplois n'accroît ni l'attractivité de métiers pénibles ni des rémunérations peu attrayantes.

Il semble d'ailleurs qu'un certain nombre de structures privées françaises développent des robots similaires, mais leur coût est un frein considérable à leur déploiement massif. Ces initiatives et expériences ne peuvent se limiter à quelques structures privées.

Le plan régional IA 2021, présenté en 2018, contient un ensemble très complet d'initiatives visant à faciliter l'usage de l'intelligence artificielle par les entreprises franciliennes, à développer la formation et à lancer des challenges pour des filières prioritaires. prioritaires. La collaboration entre les collectivités territoriales et les start-up permet d'expérimenter des solutions innovantes dans des champs très variés : sécurité, transports et mobilité, transition énergétique, aménagement, urbanisme, santé ... Je pense par exemple à la maintenance prédictive des escalators, à la modélisation du trafic routier, à la réutilisation des déchets du BTP, au calcul de trajets pour les personnes handicapées ou à la création de véritables plateformes de télémédecine, pour lutter contre les déserts médicaux ; la première d'entre elles a été inaugurée à Moigny-sur-École. Ces nouvelles réponses, reposant sur l'utilisation des données et l'automatisation, ont une incidence positive sur la qualité de vie de nos concitoyens et contribuent à l'attractivité du territoire. Or cette dynamique, particulièrement forte dans ma région, engendre des coûts importants. Il est absolument nécessaire que l'État apporte son soutien financier, d'autant que le rapport de nos collègues Marie Mercier et René-Paul Savary, que je félicite pour leur travail très approfondi, pointe la difficulté, dans notre pays, de passer de la phase de recherche à la mise en application sur le terrain et à faire des avancées technologiques permises par les chercheurs des réussites économiques.